en raison de conditions climatiques particulièrement douces qui ont provoqué l'infestation précoce de pucerons verts, vecteurs de la jaunisse virale.

Il est urgent de trouver des solutions robustes pour indemniser les betteraviers les plus touchés. Alors que les pertes financières sur la récolte 2020 sont estimées à 285 millions d'euros,

Elle cumule 700 000 euros de dettes, dont 200 000 euros de redevances dues à la municipalité. Monsieur le ministre, élus et éleveurs se battent sur le terrain pour conserver cette structure de proximité, qui permet la mise en place de circuits courts, préserve au mieux le bien-être animal et assure la sauvegarde du label « veau élevé sous la mère ». Lors de notre dernier échange, vous avez affirmé votre volonté d'accompagner les abattoirs locaux sur le plan financier, notamment pour soutenir la modernisation et accroître la rentabilité de ces outils. Forte de cette logique, la municipalité de Ribérac a déposé ces derniers jours, dans le cadre du plan de relance, un projet ambitieux de création d'une salle de découpe et de transformation sur le site, de nature à sauver la structure tout en conservant l'abattoir.

elle est d'ores et déjà en contact avec des investisseurs et des coopératives d'éleveurs. Néanmoins, monsieur le ministre, il y a urgence : ce projet ne verra jamais le jour s'il n'est pas soutenu par l'État

assurer que l'engagement de l'État interviendra rapidement, si possible dans les trois mois ? Enfin, envisagez-vous des dispositifs spécifiques pour encourager l'investissement privé dans des structures comme Ribérac

je tiens à rappeler que la chasse permet de réguler la prolifération de certaines espèces, et ainsi de protéger les futures récoltes. Il va de soi cette régulation ne peut intervenir que durant une certaine période, prenant en compte le cycle de reproduction des espèces. En d'autres termes, il ne sera pas possible d'y revenir ultérieurement.

Monsieur le ministre des outre-mer, ma question porte sur le plan de relance et sa déclinaison guyanaise. Sur les 100 milliards d'euros engagés d'ici à 2022, 1,5 milliard sont destinés aux outre-mer.

de l'ingénierie nécessaire pour les réaliser dans le délai imparti, soit avant 2022, étant donné l'ampleur actuelle de la sous-consommation ou de la sous-exécution des crédits dévolus aux outre-mer Des fonds leur seront-ils alloués pour leur donner les moyens et la possibilité d'intervenir ? Je pense en particulier à la collectivité territoriale de Guyane, dont le rebasage tarde : elle est un acteur incontournable pour ce plan de relance !

territorialisation, notamment avec le président Rodolphe Alexandre et l'ensemble des maires de la Guyane. Un premier comité régional a été installé ; il va continuer à travailler et à nous soumettre des projets. Je précise que certains crédits seront automatiques, comme ceux qui sont liés à la baisse des impôts de production, à la compensation des recettes des collectivités

Pour être relancée, il faudrait déjà que la Guyane ait atteint un certain niveau de développement. Ce n'est pas le cas, en dépit de son potentiel important dans bon nombre de secteurs : elle ne fait actuellement que vivoter, sous perfusion de transferts publics. Cessons de la mettre sous cloche, libérons l'exploitation de ses ressources de façon raisonnable et rationnelle et profitons du mouvement de différenciation qui s'annonce pour faire tomber toutes les entraves à son développement, avec des méthodes et des objectifs qui lui soient propres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par certaines intercommunalités dans l'élaboration de leur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), en particulier sur les craintes des communes membres quant à la validité validité de leur plan d'occupation des sols (POS) au 1 janvier prochain. Les communes appartenant à une intercommunalité qui s'est lancée avant le 31 décembre 2015 dans l'élaboration d'un PLUI ont pu bénéficier, à la suite de l'adoption de la loi Engagement et proximité d'une prolongation de la validité de leur plan d'occupation des sols jusqu'au 31 décembre 2020. Faute de l'adoption d'un PLUI à cette date, les POS, opposables jusque-là, seront déclarés caducs ; c'est alors le règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'appliquera dans ces communes, jusqu'à l'approbation d'un PLUI (EPCI) d'appartenance. Si le report à la fin de 2020 de la caducité des POS a octroyé aux collectivités territoriales un délai supplémentaire, il s'avère insuffisant pour les EPCI qui, au début de 2020, n'avaient pas encore achevé leurs travaux. Pour ceux-là, de nouvelles délibérations étaient nécessaires, mais la crise sanitaire intervenue dès le mois de mars a considérablement retardé les travaux des intercommunalités. Les mesures de confinement liées à la crise sanitaire, le report des élections municipales et le retard consécutif pour le renouvellement et l'installation des exécutifs intercommunaux ont perturbé la réalisation d'étapes essentielles à l'élaboration de ces PLUI.

l'application du RNU limitera considérablement leurs prérogatives en matière d'urbanisme et ne leur permettra plus d'assurer la gestion pragmatique de l'urbanisme de leur territoire. Dès lors,

toujours actifs ; ils n'étaient plus que 546 au 1 septembre 2020. Plus de 90 % des POS en vigueur ont donc été convertis en PLUI. Ainsi le nombre de communes qui reviendraient au règlement national d'urbanisme, le RNU, faute d'avoir approuvé leur PLUI s'en trouve nettement diminué.

un nouveau report n'est pas envisagé par le Gouvernement. La caducité des POS ne bloque pas les projets des collectivités. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du PLUI, le RNU permet à une collectivité d'autoriser des projets lorsque l'intérêt général le justifie et que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages en dehors de l'aire urbaine existante.

public (DSP) de l'État sont arrivées à leur terme le 31 décembre 2012 et n'ont pas été renouvelées depuis, prorogeant de fait les concessions aux conditions antérieures. Il y a un peu moins d'un an, j'avais alerté la précédente ministre de la transition écologique sur cette situation juridiquement instable de nature à porter préjudice aux collectivités du département, notamment aux communes traversées par les cours d'eau utilisés. En effet, conformément au code de l'énergie, celles-ci percevraient une redevance annuelle en cas de renouvellement de la concession notamment. Mme Borne m'avait répondu

Dans ce contexte de contentieux européen et de réflexion sur l'organisation du groupe, le Gouvernement explore la possibilité, prévue par le droit des concessions, de renouveler ces concessions sans mise en concurrence à une structure dédiée. Voilà la piste à l'étude. Le renouvellement de ces concessions, que ce soit par mise en concurrence ou une structure dédiée, s'inscrit dans une politique nationale qui vise à optimiser l'investissement dans le secteur tout en redistribuant des ressources financières aux territoires par de nouvelles redevances. Une attention particulière doit être portée au personnel de ces structures.

a besoin de disposer d'une visibilité à long terme, le personnel a besoin d'être rassuré et les collectivités locales ont besoin de projets de territoire coconstruits avec le concessionnaire. La parole

Ce projet a connu quatre Présidents de la République, dix Premiers ministres, et avec tout le respect que je vous dois, madame la secrétaire d'État, plus d'une vingtaine de ministres compétents,

a confirmé la nécessité de poursuivre à la fois le projet de stockage géologique des déchets de haute activité en couche géologique profonde, dit Cigéo, dans sa conception et dans sa réalisation, et dans sa réalisation, et les recherches sur des alternatives à cette option d'enfouissement des déchets. Dans ce contexte, le Gouvernement a souhaité que l'Andra dépose une demande de déclaration d'utilité publique. Cette dernière permettra d'engager l'instruction de l'étude d'impact du projet par les services compétents de l'État, mais également par les parties prenantes, notamment les collectivités locales. En particulier, l'Autorité environnementale aura à se prononcer sur la qualité et la complétude de cette étude. En tant que Haut-Marnaise, je n'ai que trop conscience de l'importance de ce comité de haut niveau pour les élus locaux et pour tous les acteurs et parties prenantes de ce territoire ; ce comité est un outil de concertation et de pilotage des enjeux stratégiques.

sont concernées. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté le 1 octobre 2020, les vendeurs doivent financer une étude géotechnique de conception de type G2, dont le coût est de l'ordre de 1 400 euros pour un particulier et de 900 euros pour les mairies dans le cadre d'un lotissement et par unité, et ce en sus des

que les nouvelles maisons seront construites avec des techniques adaptées pour éviter ces sinistres. La nouvelle carte nationale de l'exposition au retrait-gonflement des sols argileux a été mise à disposition sur le site

identifiées par la carte comme relevant de l'aléa faible ou comme non argileuses, entraînant une sous-estimation de l'aléa. C'était notamment le cas de la commune de Metzing, quiétait classée en zone d'aléa faible alors qu'elle a fait l'objet de deux arrêtés CatNat pour les sécheresses de 2003 et 2018. 2018. Une actualisation de la carte d'aléa était nécessaire. Elle a été menée sur la base d'une évolution des connaissances scientifiques. Le nouveau dispositif s'applique uniquement dans les zones d'exposition moyenne et forte, dans un esprit de proportionnalité et d'efficience de la réglementation. Depuis le 1 octobre 2020, une étude géotechnique est effectivement exigée lors de la vente d'un terrain, mais uniquement pour les terrains non bâtis et constructibles. Il s'agit d'une étude géotechnique de type G1, dont le coût est estimé à 500 euros,

en raison du rattrapage structurel important auquel le territoire doit faire face. Le syndicat mixte de traitement des déchets, Ileva, situé sur le territoire de trois communautés d'agglomération, a engagé toutes les procédures pour créer un outil multifilières de traitement des déchets adapté au contexte local. Ce projet d'envergure doit assurer la continuité du service en 2023 pour 528 000 habitants. Le financement lié à l'emprunt est en cours de contractualisation avec les banques. L'Agence comme condition une garantie d'emprunt des EPCI membres du syndicat mixte. Cette condition devrait s'appliquer pour les autres banques dans le cadre de la clause du. Pouvez-vous

Les EPCI ont créé le syndicat mixte pour la partie traitement et agissent dans le cadre d'un transfert de compétences, les dépenses étant financées par les contributions de ses membres. Ils subventionnent également le projet à hauteur de 40 millions d'euros, contributions d'équipements autorisées par les statuts d'Ileva. Les équipements sont réalisés dans le cadre d'une compétence obligatoire que les communautés d'agglomération continuent à exercer par le biais du syndicat mixte. En cas de dissolution du syndicat mixte, les droits et obligations sont obligatoirement transférés aux EPCI. Interrogée sur la base juridique de sa demande, l'AFD fait état d'une réponse ministérielle à une question écrite, mais celle-ci n'évoque aucun élément juridique applicable en l'état au syndicat mixte. Le principe de l'interdiction des prêts entre collectivités locales ainsi que des communes vers des groupements de communes a été réaffirmé dans une autre réponse ministérielle. Cette interdiction s'applique également du syndicat mixte vers les personnes morales qui en sont membres. Madame la secrétaire

par les communes et leurs groupements à d'autres personnes publiques. En effet, si l'article L. 2252-4 prévoit des conditions pour l'octroi de telles garanties à des personnes privées, il ne mentionne pas les personnes publiques. Par construction, il découle de cette absence de condition que les communes ont la possibilité d'octroyer des garanties d'emprunt à des personnes publiques. L'article L. 5111-4 du code prévoit que les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. Cette analyse est validée par le Comité national relatif à la fiabilité des comptes publics locaux. Le syndicat mixte de traitement des déchets Ileva a été créé par la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion, la communauté intercommunale des villes solidaires et la communauté d'agglomération du territoire de la côte Ouest, qui lui ont confié, dans l'intérêt général, la mission d'assurer le traitement et la valorisation des déchets non dangereux produits sur leur territoire. Il s'agit d'un établissement public public régi par le code général des collectivités locales. En tant que personne morale de droit public, le syndicat mixte de traitement des déchets Ileva peut bénéficier des garanties d'emprunt octroyées par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres pour faciliter la réalisation d'une opération d'intérêt public. J'ajoute que l'octroi de cette garantie par les EPCI n'emporte pas d'obligation supplémentaire par rapport au droit commun. Les contributions budgétaires au syndicat constituent en effet des dépenses obligatoires susceptibles de mandatement d'office et ont vocation à couvrir les charges du syndicat, notamment le remboursement d'éventuels emprunts.

Madame la secrétaire d'État, crise sanitaire, quatorzaine imposée unilatéralement par la Grande-Bretagne, Brexit : la filière transmanche subit une baisse de trafic considérable. Quelque 5 000 salariés et, plus largement, 12 500 emplois indirects sont en jeu.

Les compagnies qui opèrent en délégation de service public, sur la ligne Dieppe-Newhaven par exemple, en sont exclues. Cela crée une inexplicable distorsion de concurrence. Je rappelle que les deux ferries de Dieppe enregistrent une baisse de deux tiers du trafic de passagers. L'opérateur évoque des suppressions d'emplois des départs volontaires. Le directeur de la ligne et l'ensemble des élus locaux demandent l'appui de tous. L'avenir du trafic transmanche est important pour les régions concernées, en premier lieu la Normandie. La ligne Dieppe-Newhaven est empruntée

La moitié des dépenses effectuées en France par les Britanniques est liée aux passages transmanche. Il est donc nécessaire de mettre en oeuvre un plan « ferry qui aille au-delà des premières mesures évoquées. L'État doit s'engager davantage, y compris en obtenant des fonds européens, en travaillant au développement

et des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre de 75 %- ce qui est absolument colossal -par rapport à 2019. En outre, comme vous l'avez souligné, la décision britannique d'instaurer une quatorzaine en plein mois d'août à toute personne entrant au Royaume-Uni n'a pas permis à ces armateurs de réaliser une saison estivale satisfaisante. Le Gouvernement a porté dès le début de la crise une attention toute particulière aux compagnies de transport de passagers, notamment en mettant en place puis en prolongeant

mais il n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Des échanges avec les organisations syndicalessont nécessaires, mais cette mesure pourrait trouver à s'appliquer aux ferries en fonction de la tendance de reprise. Enfin, à la suite de nombreux échanges avec les armateurs, le Premier ministre a annoncé en septembre dernier le principe du remboursement pour une durée d'un an des cotisations sociales des salariés. Cet effort, d'un montant estimé entre 24 millions et 30 millions d'euros pour l'ensemble des compagnies de ferry actives sur les liaisons internationales hors délégation de service public, a été inscrit dans le

entre Fontenay-le-Comte et Rochefort afin de désengorger les routes entre la Vendée et la Charente-Maritime, notamment pendant la période estivale. L'État s'est engagé à proposer des solutions alternatives dans le cadre du contrat d'avenir. Après deux réunions au ministère, trois scénarios, dont un autoroutier, ont été présentés. Dans un courrier datant du 2 octobre dernier, le président du conseil départemental de Vendée a fait savoir au ministre que les deux solutions alternatives proposées ne pouvaient être retenues, à la fois en raison de leur impact environnemental et de leur coût, mais également au regard de l'itinéraire, qui prévoit la coupure en deux fois deux voies de la commune de L'Île-d'Elle et des conditions de passage à proximité des zones urbanisées de la commune de Vix. Le projet d'autoroute est celui qui s'impose naturellement en complément du réseau existant. La Vendée et la Charente-Maritime attendent ce projet, qui fait d'ailleurs l'objet d'un très large consensus historique, indispensable pour doter le territoire d'une infrastructure de transport à la hauteur de son dynamisme.

de réduction et de compensation des impacts. Vous le savez, la déclaration d'utilité publique est désormais caduque. Compte tenu de la nécessité d'apporter des réponses aux besoins de déplacements de la Vendée et de la Charente-Maritime, y compris au droit de la commune de Marans, l'État a proposé d'accompagner les collectivités dans un projet alternatif, moins consommateur d'espace et avec un impact environnemental moindre. Comme convenu lors d'un rendez-vous en juillet dernier entre le ministre délégué chargé des transports et les élus locaux, l'État a transmisles études réalisées en ce sens par ses services. vous l'avez souligné, le président du conseil départemental de Vendée a jugé que les alternatives proposées ne pouvaient pas être retenues, sans toutefois proposer de solution qui répondrait aux difficultés rencontrées sur le plan environnemental. Le ministre chargé des transports est par ailleurs à l'écoute des retours des autres collectivités également parties prenantes au projet. Alors que le dialogue social n'a pas été poussé jusqu'au bout et que nous devons encore explorer certaines options, il n'apparaît pas possible à ce stade de conclure que la seule issue soit le tracé A831 initial. Les services de l'État restent donc disponibles pour échanger sur les pistes et solutions alternatives, y compris sur la possibilité d'une réalisation partielle au

Je vous remercie

Madame la secrétaire d'État, le fonds de solidarité pour le logement, le FSL, accorde des aides financières à des personnes en difficulté d'accès à un logement locatif, ou qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des fournitures d'eau, d'énergie ou de services de télécommunication. Tous les départements sont désormais confrontés à la multiplication du nombre de fournisseurs d'énergie. En Isère, par exemple, un client a le choix entre trente-quatre fournisseurs d'électricité et vingt fournisseurs de gaz, différents. Parmi eux, seuls trois financent historiquement le FSL.

et d'encadrer la contribution financière au FSL de tous les fournisseurs d'énergie, d'eau ou de services de télécommunication ? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice

Ce projet prévoit notamment un quartier mixte composé de logements, d'activités économiques, et d'équipements publics, dont un groupe scolaire. Il envisage aussi, à terme, la réhabilitation et l'ouverture au public du parc du Fort, la construction d'un nouvel équipement sportif, la requalification de la route départementale D4, et la création d'une trame verte et bleue.

? Êtes-vous en mesure de préciser les prochaines modalités d'un dialogue constructif entre l'État, les Canavérois et leurs élus locaux, afin de permettre la réalisation de ce projet d'aménagement durable tant attendu par la population et encore récemment souhaité par l'État ?

finance plus de 80 000 places d'hébergement, chaque nuit, en Île-de-France, pour venir en aide aux publics les plus fragiles. Parmi ces places, 10 000 ont été créées pendant le premier confinement et déjà plus de 5 000 depuis le 17 octobre, pour faire face à la croissance des besoins. besoins. Dans le contexte de la crise sanitaire, le Gouvernement a ouvert plus de 190 000 places d'hébergement d'urgence, dont 14 000 places depuis le 17 octobre dernier et 28 000 ouvertes lors du confinement du mois de mars et qui sont actuellement maintenues. Au-delà de l'hébergement d'urgence, nous portons une politique volontariste dans le cadre du plan quinquennal pour le logement d'abord, afin de développer des solutions pérennes pour ceux de nos concitoyens qui en ont besoin. C'est la raison pour laquelle le prédécesseur d'Emmanuelle Wargon avait validé la mise en oeuvre d'une expérimentation

Il s'agit, en l'occurrence, des emprises de la voie de desserte orientale sur les communes de Chennevières-sur-Marne dans le Val-de-Marne, d'Antony dans les Hauts-de-Seine et d'Éragny-sur-Oise dans le Val-d'Oise. Le Gouvernement est attaché à la concertation,

qui montrent qu'il est possible de développer à la fois une solution technique innovante, une trajectoire économique équilibrée et un projet social adapté à la réalité de ces trois communes.

et de la relance. Monsieur le secrétaire d'État, lorsqu'un assuré titulaire d'une assurance vie opte pour une sortie de son contrat sous la forme d'une rente, on parle alors de rente viagère.

La part imposable varie avec l'âge du bénéficiaire : à titre d'exemple, la fraction imposable est de 40 %, si le crédirentier est âgé de 60 à 69 ans, lors de l'entrée en jouissance de la rente.

La base de calcul qui a servi à établir la part imposable des rentes viagères se fonde sur le taux d'intérêt technique, c'est-à-dire le taux que l'assureur prend en compte dans la modélisation du risque qu'il s'apprête à couvrir, en vue d'établir la tarification du contrat. Cependant, le taux d'intérêt retenu pour la fiscalité des rentes viagères, à 3,50

Face à cette situation injuste, il est indispensable de réformer la fiscalité des rentes viagères, afin de calculer l'impôt en fonction du revenu réellement imposable.

qui accepte de se dessaisir d'un élément de son patrimoine, immobilier ou mobilier, en contrepartie de versements effectués à son profit sa vie durant. Ces versements, appelés « arrérages », correspondent pour partie au remboursement du capital aliéné et pour partie à la rémunération de ce capital. Conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, les RVTO ne sont imposables que pour une fraction de leur montant décroissante en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. vous l'avez rappelé, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 %, selon que le crédirentier est alors âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d'au moins 70 ans. Cette fraction taxable correspond aux arrérages représentatifs des seuls intérêts produits par le capital aliéné. Ainsi, le système actuel de taxation des RVTO est économiquement justifié. Il permet d'exclure du champ de l'impôt sur le revenu la part de la rente réputée couvrir le remboursement du capital. Le fait que la fraction imposable de la rente soit déterminée de manière forfaitaire peut certes conduire à s'écarter de la répartition effective entre remboursement du capital aliéné et rémunération de ce capital, à un moment donné au cours de la période de versement de la rente. Toutefois, l'écart peut aussi apparaître, à l'inverse, au profit du crédirentier, et l'équilibre doit s'apprécier sur la durée, potentiellement longue, de versement de la rente. En outre, ce barème forfaitaire présente l'avantage d'être simple à appliquer et équitable dans la mesure où plus l'assuré est âgé lors de l'aliénation de son capital, moins la fraction imposée de la rente est élevée, dès lors que, en moyenne, la part des intérêts dans la rente est inférieure. Au demeurant, une réforme du régime d'imposition des RVTO motivée par l'évolution des taux d'intérêt, par nature conjoncturelle, risquerait de conduire à sa révision permanente et de compromettre sa lisibilité et sa prévisibilité pour les épargnants,

qui ont la garde de leurs enfants à la suite d'une séparation. La monoparentalité pose des difficultés d'organisation et entraîne une baisse notable du niveau de vie. Près de quatre familles monoparentales sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 2,8 millions d'enfants sont en situation de pauvreté ; 85 % des familles monoparentales ont à leur tête une femme. une femme. La pension alimentaire, versée en cas de divorce ou de séparation de corps, en vertu de l'article 373-2-2 du code civil, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire prévu à l'article 373-2-4 sont déductibles du revenu global de la personne qui verse la pension, mais constituent un revenu imposable entre les mains de la bénéficiaire. de la bénéficiaire. Afin de lutter contre la pauvreté des familles monoparentales, je souhaiterais savoir- si possible, avant ma retraite une réflexion sur la déductibilité fiscale de la pension alimentaire pour son bénéficiaire, dans la limite d'un certain plafond. La parole est à M. le secrétaire

la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la CEEE, prévue par L'article 373-2-2 du code civil ainsi que son complément prévu à l'article 373-2-4 du code civil prennent la forme, dans les faits, d'une pension alimentaire. En application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le débiteur de la pension peut la déduire de son revenu imposable dès lors qu'elle est effectivement versée. Il importe toutefois que le ou les enfants mineurs pour lesquels la pension alimentaire est est versée ne soient pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial, afin de ne pas octroyer un double avantage pour le parent qui verse la pension : majoration du quotient familial et réduction du revenu imposable. En application des articles 12 et 79 du CGI, les pensions alimentaires sont corrélativement imposables chez le parent bénéficiaire, à condition qu'il les ait effectivement perçues. Dans le cas particulier de la garde alternée, la charge d'entretien des enfants est présumée partagée entre les parents. Les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit- majorations du quotient, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux -sont en conséquence répartis par moitié entre les ex-conjoints. Les contribuables ne peuvent alors opérer aucune déduction au titre des pensions alimentaires versées pour leurs enfants mineurs, dès lors que ceux-ci sont pris en compte pour la détermination de leur quotient familial. Corrélativement, les pensions alimentaires ainsi versées ne sont, dans ce cas, pas imposables au nom de leur bénéficiaire. Toutefois, s'il apparaît que l'un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires versées par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux. Dans cette situation, l'autre parent peut alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement, cette pension étant alors imposable chez celui qui la reçoit. En outre, l'impôt sur le revenu prend en compte d'une autre manière la situation particulière des familles monoparentales les contribuables qui vivent seuls et supportent effectivement la charge principale ou exclusive de leurs enfants bénéficient ainsi d'une part entière de quotient familial pour le premier d'entre eux, l'avantage maximal en impôt procuré par cette part étant fixé, pour 2019, à 3 697 euros. Enfin, la fiscalité n'est pas le seul moyen de venir en aide aux familles monoparentales. Il existe plusieurs aides sociales qui participent de cet objectif, notamment les allocations familiales, le complément familial versé sous condition de ressources aux parents isolés ayant au moins trois enfants, l'allocation de soutien familial, l'ASF, qui est versée aux personnes qui élèvent seules leur enfant privé de l'aide de l'un de ses parents, ou bien pour compléter une pension alimentaire dont le montant est faible. Ces prestations familiales ne sont pas imposables. Dès lors, le Gouvernement n'est pas favorable à une modification du régime d'imposition des pensions alimentaires. La parole est à Mme Michelle Gréaume, auteure de la question

de la relance. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Vallourec a confirmé un plan de 1 000 nouvelles suppressions d'emplois dont 350 en France, 190 à Déville-lès-Rouen dont le site sera fermé, 30 au siège social et 130 dans le département du Nord, où l'avenir des de Valenciennes, Aulnoye-Aymeries et Saint-Saulve est des plus sombres. Les syndicats salariés alertent depuis longtemps sur les risques d'un nouveau plan social, et sollicitent l'intervention urgente de l'État, actionnaire de référence de Vallourec, à hauteur de 15 %, afin que d'autres solutions émergent. En vain ! Monsieur le secrétaire d'État, qu'avez-vous fait pour empêcher ce nouveau coup porté à l'emploi et pour préserver, malgré les difficultés, un groupe et un savoir-faire essentiels à notre souveraineté et à la transition écologique ? J'entends bien les arguments que l'on nous oppose, la dette et les intérêts qui plombent l'entreprise, le ralentissement du marché aggravé par la crise de la covid-19. Cependant, n'est-il pas temps de remettre en cause la stratégie industrielle et financière du groupe ? Choix obstiné du tout-pétrole, désinvestissement sur le territoire national, délocalisations, razzia sur les fonds publics, recherche du profit maximal, la recette est toujours la même ! Les conséquences ne varient pas non plus. Des milliers d'emplois directs et indirects sont détruits. La filière est en sous-capacité de production, ce qui place la France en position de vulnérabilité inquiétante.

ou de fonds d'investissement étrangers. La conversion de leurs créances en capital va permettre à ces groupes de faire main basse sur Vallourec et d'imposer encore plus facilement leurs conditions et leurs exigences de rentabilité. Comment peut-on les laisser faire ? Il est urgent de sortir Vallourec des griffes de la finance. Pour cela, j'avance deux propositions. Premièrement, il faut exiger des établissements financiers français qu'ils renoncent aux intérêts prélevés sur les résultats du groupe Vallourec.

Elle a subi une très forte baisse de son activité pétrolière, son principal débouché, qui pèse plus de 70 % de son chiffre d'affaires, dans un contexte mondial de contraction de l'activité d'exploration et de production. Les efforts de reconquête de la performance industrielle de Vallourec, mis en place depuis 2015, se rapprochaient des objectifs escomptés pour restaurer la compétitivité de l'activité, d'être percutés de plein fouet par la crise. L'ensemble de l'activité du groupe, à l'échelle mondiale, est désormais touché. L'entreprise a donc décidé d'entreprendre une restructuration de son outil industriel, au niveau mondial, dont les conséquences sont lourdes. Un tiers des emplois, soit 900 d'entre eux, ont été supprimés aux États-Unis, en avril dernier.

Nous menons des discussions avec les représentants syndicaux et les élus du territoire, car c'est ensemble que nous trouverons les solutions. Ma collègue Élisabeth Borne est également très mobilisée pour permettre aux salariés de bénéficier des conditions les plus protectrices possible, dans le cadre du PSE, sur l'ensemble des sites de Vallourec. Le préfet de Seine-Maritime a immédiatement réactivé le comité industriel territorial pour réfléchir aux solutions d'avenir du site. Nous savons pouvoir compter sur la mobilisation des présidents de la région Normandie et de la métropole de Rouen pour oeuvrer, ensemble, à l'implantation de nouvelles activités sur le site. Dans le Valenciennois, où 1 222 salariés travaillent sur les différents sites, ce sont 137 emplois

je sais pouvoir compter sur la mobilisation d'Élisabeth Borne, en liaison étroite avec le président de région, Xavier Bertrand, et les élus locaux. Soyez-en assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes mobilisés avec la même énergie, et notre action, aussi bien dans le Nord qu'en Seine-Maritime est guidée par la même boussole : celle de l'emploi et l'activité industrielle.

rencontrent des difficultés pour mettre en place la généralisation de l'offre de paiement en ligne. Le décret n° 2018-689 du 1 août 2018 prévoit une obligation de mise à disposition à titre gratuit par les administrations publiques d'un service de paiement en ligne à destination de leurs usagers, qu'ils soient particuliers ou entreprises.

Face à l'ampleur de la tâche, les équipes municipales ont besoin d'un contexte plus serein. Par ailleurs, tous les citoyens n'ont pas les moyens de payer en ligne. Certaines familles, en proie à des difficultés majeures, préfèrent payer directement les services de la collectivité. Dans la mesure où la France projette de développer une administration 100 % numérique d'ici à 2022, il convient de faciliter, pour tous, le recours aux outils informatiques. Comment envisagez-vous cette évolution pour les populations précarisées ? Quels moyens prévoyez-vous pour les intégrer à cette réforme de l'administration ?

L'obligation d'offre de paiement en ligne, prévue par l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2017 et le décret que vous citez, répond aux attentes des usagers, dont beaucoup plébiscitent le recours à des moyens de paiement dématérialisés, diversifiés et accessibles à toute heure et à distance. Le paiement par internet aux collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une ouverture vers la dématérialisation. La crise sanitaire actuelle a démontré la nécessité d'offrir aux usagers des moyens de paiement â distance, pour ceux qui ont un accès à internet. Il est donc important de poursuivre, voire d'accélérer, les actions permettant de satisfaire à cette obligation et, par là même, aux besoins des usagers. Il s'agit d'un intérêt partagé par les ménages comme par les collectivités, qui voient ainsi leurs recettes rentrer mieux et plus vite. Le Conseil national de l'évaluation des normes, composé de représentants des associations d'élus, ne s'y est pas trompé en donnant un avis favorable au décret. La direction générale des finances publiques, la DGFiP, est pleinement mobilisée pour accompagner les collectivités dans la mise en place d'une offre de paiement en ligne et pour aider celles qui sont en retard par rapport aux échéances du décret. Grâce à l'outil PayFiP, le paiement des sommes dues pour l'usage des services publics d'une collectivité est facilité.

besoin des usagers et participe dans le même temps à la promotion de l'administration numérique.

la France, hier encore quatrième puissance mondiale, se voit désormais rétrogradée à la sixième place ! Contre toute attente, son économie donne toutes les apparences d'un déclin que rien ne semble pouvoir enrayer. Comment est-ce possible ? Comment en est-on arrivé là ? Qui sont les responsables d'une telle situation ? Est-il juste d'incriminer les politiques pour des choix, il est vrai, parfois bien hasardeux

La liste est longue, et le maillage industriel de la France témoigne de cette vitalité économique dans des domaines très variés. Cette diversification nous permet d'affronter les crises qui secouent de façon récurrente l'économie mondiale. Pourtant, les chiffres de la paupérisation de notre pays

sur un plan davantage sémantique, ne devrait-on pas plutôt parler de « survie » ? Le ministre de l'économie, de par ses fonctions, est le plus au fait de la situation. Les élus, de par leurs mandats, y sont directement confrontés. La pauvreté est leur lot quotidien avec des permanences

la psychologie est partie prenante de l'économie. Mais comment redonner espoir et confiance dans la vie à des êtres brisés par les épreuves ? Le message répété à l'envi, qui encourage la consommation et non l'épargne, car, dites-vous, « la consommation, ce sont des emplois », est-il seulement audible ? Que peut bien consommer un smicard avec le peu qu'il a, sinon des produits à bas coût ? Votre rhétorique, il faut le reconnaître, est de grande qualité. Hélas, un discours, si bon soit-il, ne se mange pas : « je vis de bonne soupe, et non de beau langage » disait en son temps Molière. Combien avait-il raison

? La parole est à M. le secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Jean-Marie Mizzon, nous sommes d'accord sur un point : le tissu productif français est de qualité, et la France a tous les atouts pour réussir. Elle l'a prouvé, car, avant la crise, nous étions déjà en train de réussir. Je rappelle que, en 2019, notre pays était le plus attractif d'Europe pour

Avant la crise, la pauvreté reculait : en 2019, 210 000 personnes sont sorties de la pauvreté, et les inégalités de revenus se sont réduites. Le revenu médian des Français a augmenté plus vite que la croissance, notamment grâce à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et à l'exonération de charges sur les heures supplémentaires.

à la complémentaire de santé solidaire, ou la limitation des frais bancaires pour les personnes précaires. Aujourd'hui, ces précaires sont les premières victimes de la crise sanitaire et sociale. Le Gouvernement a répondu présent avec une préoccupation constante : ne laisser personne au bord du chemin. Nous avons donc pris un ensemble de mesures sociales d'urgence, afin de les aider et de prévenir l'entrée dans la pauvreté, dans des proportions jamais connues dans l'histoire de notre pays : au total, plus de 3,5 milliards d'euros d'aides directes ont été versés depuis le début de la crise.

S'agissant enfin des jeunes, le plan « Un jeune, une solution », qui est partie intégrante du plan de relance, a été annoncé en juillet dernier pour soutenir l'insertion, l'apprentissage et l'emploi des jeunes dès cet été et la rentrée. Trois mois après son lancement, nous avons déjà de premiers résultats encourageants.

l'économie numérique française continuera à se développer en 2020, plus qu'en 2019. Le numérique est déjà le secteur qui crée le plus d'emplois en France. Pour la première fois cette année, notre pays dépassera l'Allemagne en ce qui concerne la croissance de son écosystème numérique. C'est la meilleure manière de préparer l'avenir et, dans le cadre du plan de relance, cela mobilise tous nos efforts.

Ainsi, les subventions octroyées à ces structures ont considérablement baissé, pour inciter les travailleurs en situation de handicap à rejoindre les entreprises dites « ordinaires ». Or ces personnes, qui ont parfois des difficultés psychiques ou intellectuelles, peinent à trouver un emploi en milieu ordinaire, phénomène considérablement accentué par la crise que nous vivons. Les professionnels du secteur des entreprises adaptées souhaitent enfin

Les membres de l'association Action collective en faveur des entreprises adaptées insistent aussi sur la nécessité de revenir sur la disposition qui prévoit, à l'horizon de 2022, de limiter à 75 % le pourcentage de salariés handicapés dans les entreprises adaptées.

comme le CDD dit « tremplin », par exemple. Madame la secrétaire d'État, entendez-vous enfin soutenir les actions si précieuses des entreprises adaptées, en particulier dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique ? La parole

tout en développant leur dimension inclusive. Cette évolution est une nécessité si l'on veut renforcer la capacité des entreprises adaptées à proposer des parcours dynamiques d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, à répondre aux besoins de des entreprises dites « classiques

La question de fond est plutôt celle de l'évolution du positionnement des entreprises adaptées. L'emploi en milieu classique doit être recherché : nul n'est inemployable, dès lors qu'un accompagnement adapté du salarié

Un appel d'offres de 868 millions d'euros a déjà été lancé, et beaucoup d'entreprises adaptées y ont répondu. Le comité scientifique d'évaluation de la réforme prévue par la loi de 2009 sera lancé d'ici la fin de l'année : il permettra d'évaluer l'impact de cette évolution, à laquelle adhère pleinement l'Union nationale des entreprises adaptées,

Nous sommes à leurs côtés, et nous le resterons.

Madame la présidente, comme vous l'indiquez, ma question s'adresse à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, et concerne l'absence de renouvellement des membres de la commission du droit local d'Alsace-Moselle.

était de répondre à la très forte attente des Alsaciens de voir leurs spécificités locales prises en compte. Chargée d'étudier et de proposer toute mesure « relative au droit particulier applicable dans les trois départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin », cette commission mérite incontestablement de continuer à oeuvrer, car, comme vous le savez peut-être, selon les sondages, 80 % à 90 % des Alsaciens se disent attachés à leur droit local. Or, faute de nomination, le mandat de ses membres ayant pris fin il y a près d'un an et demi maintenant, la commission du droit local d'Alsace-Moselle n'est plus autorisée statutairement

À quatre semaines de la mise en place de la collectivité européenne d'Alsace, les Alsaciens ne comprendraient pas que cette instance n'existe pas. Ce serait naturellement un coup très dur porté à l'Alsace naissante. Je vous remercie des précisions que vous voudrez bien apporter sur

Il résulte en effet des dispositions de l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration que les commissions administratives consultatives créées par décret le sont pour une durée maximale de cinq ans. L'absence d'existence légale de la commission fait donc obstacle à la nomination de nouveaux membres. Conformément à la circulaire du 12 septembre 2018 du Premier ministre Édouard Philippe relative à la réduction du nombre des commissions consultatives, une reprise d'activité de la commission, qui serait en réalité analysée comme la création d'une nouvelle commission, devrait normalement être précédée de la suppression de deux autres commissions consultatives. Le Gouvernement étant cependant particulièrement sensible aux spécificités et à la richesse du droit local d'Alsace-Moselle, qui bénéficie par ailleurs de l'expertise de l'Institut du droit local alsacien-mosellan, ministre de la justice est tout disposé à travailler à la meilleure façon de les prendre en compte, en étroite concertation avec les élus et les représentants des trois départements concernés, et ce dans un cadre qui reste à définir.

refusent toujours de pratiquer des IVG, en invoquant la clause de conscience, mais le manque de médecins et de sages-femmes dans certains territoires, qui sont de véritables déserts médicaux, et les fermetures de services éloignent de toute solution les femmes souhaitant y avoir recours.

Pourtant, les déserts médicaux subsistent, et l'accompagnement sur les questions liées à la vie sexuelle et contraceptive est encore limité ou peu accessible. Or toutes les femmes, quels que soient leurs ressources ou leur lieu d'habitation, doivent pouvoir recourir à une IVG et bénéficier d'un accompagnement si elles le veulent. Il s'agit là d'une question de justice et d'égalité. C'est pourquoi je souhaite connaître les mesures et initiatives que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour favoriser un égal accès à l'information et aux moyens de contraception, qui ne sont toujours

À cet égard, le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes collabore de façon étroite avec le ministère des solidarités et de la santé, qui pilote cette politique publique. Le Gouvernement a mis en place de nombreuses dispositions pendant la crise sanitaire, pour maintenir l'accès des femmes à l'IVG et favoriser les IVG en ville, comme la promotion de la téléconsultation et l'allongement de deux semaines du délai des IVG médicamenteuses en ville, ce qui a bénéficié aux territoires en tension, comme les Hauts-de-France. mesures, le Gouvernement a annoncé à la fin de 2019 un ensemble de dispositifs qui sont en cours de déploiement : l'inscription de l'IVG comme action prioritaire de la formation continue des médecins et des sages-femmes, la mise en place d'un annuaire exhaustif et actualisé de l'offre d'IVG dans chaque région, ciblés par les agences régionales de santé, les ARS, et ce de façon systématique lorsque des territoires en tension sont identifiés. Les taux de recours à l'IVG connaissent de fortes variations selon les territoires. Ils sont plus élevés dans les territoires d'outre-mer, en Île-de-France et dans le Sud-Est.

Concernant la situation particulière des Hauts-de-France, le délai d'accès à l'IVG montre que cette région se situe parmi les huit qui déclarent des délais moyens supérieurs à huit jours.

Par ailleurs, j'attends de vous et de vos collègues, en particulier de Mme Elisabeth Moreno, que vous vérifiez que ce maillage territorial, sur lequel je vous interrogeais, soit vraiment susceptible d'apporter des réponses à toutes les femmes et dans tous les territoires, car je me permets d'insister : ce n'est pas le cas dans les Hauts-de-France. Dans certaines zones de mon département, il y a encore beaucoup de travail

Madame la ministre, j'appelle votre attention sur l'enjeu lié au diagnostic et à la prise en charge précoce du sepsis, autrement dit d'une septicémie, complication la plus grave des infections. Le sepsis touche chaque année environ 30 millions de personnes et entraîne 6 millions de décès de décès dans le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. On compte en France au moins 180 000 personnes, de tout âge, victimes d'un sepsis chaque année. La mortalité est de 27 % et peut atteindre 50 % dans sa forme la plus sévère, que l'on appelle le choc septique. de la première cause de mortalité en service de réanimation et de l'une des premières causes de mortalité intrahospitalière. Face à ces chiffres, les autorités, les spécialistes et les sociétés concernés se sont mobilisés.

La gravité est souvent liée à un diagnostic tardif et à une hétérogénéité dans la prise en charge des patients. La précocité du diagnostic et un protocole de soins adapté sont donc au coeur des travaux. La délocalisation du diagnostic au plus près du patient, au sein des services d'urgence notamment, ainsi que l'élaboration d'un protocole national de prise en charge, adaptée du référentiel international de la, apparaissent dès lors comme des pistes à considérer.

en place les préconisations du rapport du professeur Djillali Annane et des sociétés savantes sont bien avancés. Les recommandations relatives à l'amélioration du parcours de soins que vous évoquez sont en cours de rédaction

Si certains travaux ont pu connaître du retard en raison de la crise sanitaire actuelle, la recherche sur le sepsis a, quant à elle, bénéficié d'un intérêt approfondi, puisque, comme vous le savez, cette maladie est l'une des complications majeures de la covid-19. De nombreux essais cliniques sur des molécules immuno-modulatrices sont en cours, et des appels à projets de Bpifrance pour l'amélioration du diagnostic du sepsis ont été lancés. La France avance donc à grands pas, madame la sénatrice. Toujours en termes de recherche, le projet Sepsis porté par Djillali Annane figure parmi les vingt et un nouveaux lauréats de l'appel à projets Fédérations hospitalo-universitaires, ou FHU, qui a été annoncé en décembre 2019 et que vous évoquiez. Une plateforme épidémiologique nationale a par ailleurs été mise en place, ce qui permettra d'améliorer les connaissances sur les incidences du sepsis, ses caractéristiques et le suivi de son évolution. Concomitamment, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, en lien avec la direction générale de la santé et les sociétés savantes, vient de finaliser la révision du fascicule de codage des pathologies infectieuses pour le programme de médicalisation des systèmes d'information. Ce document comporte de nouvelles consignes de codage du sepsis et sera diffusé auprès des professionnels de santé dès le début de l'année prochaine.

ces préconisations puissent trouver très rapidement une issue pour traiter cette maladie, qui touche de nombreux patients et qui a des conséquences souvent dramatiques.

et de la santé. Madame la ministre, ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités et de la santé et porte sur les difficultés rencontrées par les établissements de santé privés d'intérêt collectif, tout particulièrement le centre hospitalier Sainte-Marie en Haute-Loire. En effet, cet établissement fait partie d'une association à but non lucratif, qui est la seule structure du département à assurer des missions de service public en psychiatrie pour les enfants et les adultes. La pénurie de professionnels de santé met en péril l'activité et la capacité de cet établissement à exercer ses missions. Les principales inquiétudes concernent bien sûr les praticiens en poste, mais également les recrutements. La pyramide des âges de cette structure devient inquiétante, avec au moins deux tiers de médecins âgés de plus de 50 ans : c'est un signal d'alerte fort. Les écarts de rémunération, qui se creusent entre les grilles de la convention collective du 31 octobre 1951 et celle des praticiens hospitaliers, constituent en outre un obstacle à l'embauche. La suppression des trois premiers échelons de la grille des salaires des praticiens hospitaliers, décidée récemment, ne fait que renforcer cette inégalité. C'est pourquoi le recours à l'intérim devient aujourd'hui inévitable de garantir la continuité des soins, mais cette option n'est absolument pas une solution durable, en raison de son coût élevé et de compétences parfois peu conformes à celles qui D'autres obstacles propres au statut des établissements privés viennent s'ajouter à ceux que je viens de mentionner : la non-reconnaissance de l'exercice en établissement de santé privé pour le concours de praticien hospitalier, la quasi-impossibilité d'obtenir le détachement d'un centre hospitalier public vers ces établissements et, enfin, la faible attractivité du territoire. Enfin, les établissements de santé privés, tels que le centre Sainte-Marie,

À l'image du Ségur de la santé ou de l'attribution des primes exceptionnelles dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, cette situation montre une nouvelle fois une distinction clivante entre les établissements sous statut public et les établissements sous statut privé. Madame la ministre, je souhaiterais connaître votre position sur la place qui est réellement accordée aux établissements de santé privés d'intérêt collectif. Pourquoi ces derniers ne peuvent-ils pas bénéficier des mêmes autorisations en termes de recrutement

Comme vous le savez, notre système hospitalier repose sur plusieurs modèles d'établissement : le public, le privé, le non lucratif et le privé lucratif. L'action du Gouvernement vise à favoriser la coopération et la complémentarité

rappeler que les Espic bénéficieront très largement du Ségur de la santé, que ce soit la revalorisation des sages-femmes et des personnels non médicaux, le plan d'investissement ou encore la réforme du troisième cycle des études de médecine, qui ouvre la possibilité de réaliser des stages dans ces établissements, et accroît en conséquence leur attractivité. Par ailleurs, comme vous le savez, les Espic bénéficient d'une certaine souplesse en matière d'embauche et de rémunération des médecins dans le cadre de leur convention collective, liberté que le statut n'offre pas aux établissements publics, dans lesquels des grilles encadrent les rémunérations des praticiens hospitaliers.

l'exercice mixte des praticiens entre secteur public et secteur privé. Les textes d'application de cette mesure seront prochainement publiés et auront un effet sur l'attractivité des carrières, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Soyez assuré que le Gouvernement est attentif à la situation, à l'attractivité des Espic et à la reconnaissance de leur légitime place au coeur du système de santé français. Loin du clivage que vous évoquez, nous entretenons avec les représentants de ces établissements des relations étroites et constructives. Ils ont d'ailleurs engagé des discussions avec les fédérations représentatives des établissements de santé privés, afin d'objectiver un éventuel différentiel d'attractivité entre secteur public et secteur privé, en tenant compte, bien sûr, de l'impact du Ségur de la santé.

C'est une charge qui ne cesse de s'alourdir, compte tenu de la revalorisation du montant de l'allocation décidée par l'État entre 2013 et 2017, et de l'augmentation constante du nombre de bénéficiaires depuis 2010. J'ajoute que la crise économique est en train de jeter dans la pauvreté un nombre considérable de ménages et que les départements seront naturellement en première ligne pour assurer la solidarité nécessaire. Plus que l'augmentation du nombre d'allocataires du RSA, c'est la compensation très insuffisante de l'État qui fragilise la situation financière des départements. Dans ce contexte très incertain, l'accentuation de la lutte contre la fraude s'avère indispensable. À titre d'exemple, dans mon département, l'Essonne, plusieurs actions pour détecter et sanctionner les actes délibérés d'omission de déclaration ou de fausse déclaration ont été mises en oeuvre. Le conseil départemental a notamment instauré des amendes administratives et créé un service de contrôle des données. Le partage d'informations avec la caisse d'allocations familiales et Pôle emploi contribue également à rendre plus efficace la lutte contre la fraude. Néanmoins, il faut aller plus loin Le Gouvernement est-il prêt à donner aux départements la possibilité d'accéder au Fichier national des comptes bancaires et assimilés, le Ficoba, afin d'obtenir la liste des comptes des allocataires faisant l'objet d'un contrôle- il me semble important de souligner que le RSA est la seule allocation susceptible d'être versée sur le compte d'un tiers Est-il prêt à leur octroyer la faculté de mener des contrôles des ouvertures de droit au RSA ? Est-il prêt, enfin, à leur permettre d'accéder à certaines informations du répertoire national commun de la protection sociale,

que de situations de recours abusifs aux aides sociales. C'est pourquoi, depuis le début des années 2010, les branches de régime général de la sécurité sociale et Pôle emploi détectent et sanctionnent les cas de fraude, parfois pour des montants élevés- pour un nombre croissant d'entre elles, d'ailleurs, l'intentionnalité de l'auteur de l'irrégularité n'est pas démontrée. La branche famille, compétente en matière de contrôle s'agissant du RSA, a détecté 323,7 millions d'euros d'euros de préjudices subis au titre des fraudes en 2019, soit 3,6 fois plus qu'en 2010. À lui seul, le RSA a représenté à peu près 46 % des fautes qualifiées en 2019. L'omission et les fausses déclarations de ressources constituent le premier mode opératoire des fraudes et fautes détectées. Les organismes sociaux mènent des actions de contrôle, mais peuvent également prévenir la fraude en agissant. Pour autant, la Cour des comptes, dans son rapport sur la lutte contre les fraudes, a relevé que les erreurs déclaratives des allocataires des caisses d'allocations familiales étaient la principale origine des trop-perçus de prestations. Le RSA et la prime d'activité figurent parmi les principales prestations affectées par ces erreurs. La mise en place du dispositif de ressources mensuelles, regroupant la très grande majorité des données relatives aux ressources- revenus d'activité, prestations sociales, revenus du capital -permet de limiter les erreurs, volontaires ou non, par l'échange d'informations entre les sphères sociale et fiscale, à la suite de la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. De nombreuses mesures sont d'ores et déjà mises en oeuvre, pour agir efficacement contre la fraude au RSA.

face aux difficultés exceptionnelles auxquelles sont confrontés les départements, leur baisse de recettes et l'augmentation des demandes, l'État leur proposera une expérimentation de recentralisation du financement du RSA.

a mis en place un parcours de soins global après le traitement d'un cancer. Ce parcours de soins vise à améliorer la prise en charge des personnes malades, en leur proposant un accès systématique à des soins de support, notamment à des activités physiques et sportives. Il comprend spécifiquement la prise en charge d'un bilan d'activité physique pouvant, par la suite, déboucher sur une prescription d'activité physique, comme le prévoit l'article 144 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. À ce jour, aucun décret d'application n'a été publié, ce qui ne permet pas de mettre en place ces parcours et de déployer la prescription d'activité physique, dont les effets sont pourtant indéniables sur la santé. C'est regrettable. Les effets de l'activité physique thérapeutique sont largement prouvés ; il est urgent que notre système de santé y ait recours. Les bénéfices, tant en termes médicaux qu'en termes économiques, ne sont plus à démontrer.

Enfin, une fois ces bilans réalisés, les patients atteints du cancer devront être orientés. C'est pourquoi il faut encourager largement ces pratiques et renforcer la formation et l'information des professionnels. Il est urgent d'accompagner les patients, mais également les professionnels de santé. Aussi, pourriez-vous m'indiquer votre calendrier sur ce dispositif, mais également vos intentions pour soutenir et développer le sport sur ordonnance en France ?

voilà quelques années. Plus de 3 millions de personnes vivent aujourd'hui en France avec un cancer. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année augmente, les progrès réalisés dans le diagnostic et les traitements ont permis de faire reculer la mortalité. Être atteint d'un cancer demeure une épreuve, bien sûr, pour les patients et ceux qui leur sont chers. L'intérêt des soins de support en post-traitement sur la qualité de vie, notamment l'activité physique dont vous parlez, n'est plus à démontrer. C'est pourquoi le Gouvernement a souhaité mettre en place un parcours d'accompagnement vers l'après-cancer, introduit à l'article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce dispositif vise à améliorer la prise en charge des personnes malades, en proposant sur prescription, en fonction des besoins du patient, jusqu'à une année après le traitement et pendant un an, différentes consultations visant à dresser un bilan d'activité physique, psychologique nutritionnel, voire des consultations sur plusieurs de ces plans, notamment psychologiques.

La publication des textes réglementaires et des instructions associées se fera pratiquement en simultané, soit avant la fin de l'année. En conséquence, la mise en oeuvre du parcours pourrait se faire entre la fin d'année et le début d'année prochaine. Les ARS seront chargées de sélectionner les structures qui proposeront ces parcours et devront établir une convention avec elles, afin de permettre leur financement. Ce parcours post-cancer illustre notre volonté de développer le sport sur ordonnance, en permettant une prise en charge à 100 % des bilans d'activité physique adaptée et des soins de support. Ce dispositif devrait faciliter la transition entre hôpital et ville, tout en améliorant la qualité de vie des patients.

Par ailleurs, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit une expérimentation similaire pour les personnes atteintes de diabète et d'hypertension artérielle. Espérons que la mise en oeuvre sera beaucoup plus rapide pour ces pathologies

pour les établissements de santé et pour les Ehpad, la question des établissements sociaux et médico-sociaux a également été abordée. S'agissant des revalorisations salariales d'ores et déjà souhaitées, un temps d'expertise complémentaire a été jugé nécessaire pour faire la lumière sur des situations qui- vous le dites vous-même

relevant de différents financeurs. Ne faisons pas semblant de croire que le sujet est simple à aborder et à régler ! Ce travail, qui était prévu par les accords du Ségur de la santé, Après une première rencontre avec les partenaires sociaux de la fonction publique hospitalière, une organisation est en train d'être posée pour aboutir rapidement. Le Gouvernement a demandé à Michel Laforcade,

pour nous, le libre choix du lieu de résidence- en établissement ou à domicile -doit être particulièrement respecté. Il serait préjudiciable que les personnels intervenant auprès de ceux qui ont fait le choix de rester à domicile soient pénalisés financièrement par rapport à ceux qui travaillent en institution.

Le service de santé des armées a vu, ces dernières années, une politique de réduction de ses coûts, avec, notamment, la fermeture de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris. En Gironde, c'est l'hôpital Robert-Picqué, situé à Villenave-d'Ornon, dont la fermeture est programmée pour 2021. L'hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué accueille 80 % de civils. Il est reconnu pour la compétence de son personnel et la qualité des soins. Il dispose d'une situation privilégiée, d'un accès facile et dessert toute la zone sud de la métropole bordelaise, soit un bassin de vie de près de 200 000 personnes. Il traite 28 000 urgences par an et possède 242 lits d'hospitalisation. Cet hôpital, rénové en 2001, dispose des différentes certifications et accréditations de qualité pour continuer à fonctionner. Il est également l'un des rares établissements ayant encore une structure pavillonnaire pour prendre en charge, dans de bonnes conditions, les patients infectés. Il est en outre doté d'un héliport, qui ne pourrait être transféré nulle part ailleurs. L'hôpital Robert-Picqué a rendu de grands services lors de la première vague de l'épidémie. En augmentant sa capacité d'accueil de 10 à 15 lits en réanimation, il a pu accueillir une dizaine de patients du Grand Est. L'hôpital est plus que jamais actif lors de cette deuxième vague, avec ses services de soins, notamment les urgences, et la réanimation. Je vous demande donc, madame la ministre, que soit réétudié le transfert de ses activités pour répondre à la crise sanitaire actuelle, ainsi qu'aux futures pandémies,

je vous remercie tout d'abord des paroles que vous avez eues pour les médecins et personnels de l'hôpital Robert-Picqué, qui, effectivement, ont réalisé un important travail dans cette crise sanitaire.

faire en sorte que le service de santé des armées soit essentiellement tourné vers le soutien aux forces armées, ce qui est sa mission prioritaire, pour répondre aux contrats opérationnels de nos armées et, bien sûr, poursuivre la montée en compétences de ses médecins, de ses infirmiers et de tous ses personnels, afin que ceux-ci puissent également répondre à ces objectifs opérationnels. Le rapprochement des hôpitaux, notamment Robert-Picqué, avec la santé publique vise, lui aussi, des objectifs très précis. Il s'agit d'améliorer l'offre de soins sur le territoire

les économies demandées, chaque année, par Bercy. Ainsi, 231 postes ont été supprimés entre 2018 et 2020. Le Gouvernement a annoncé l'arrêt de l'hémorragie pour 2021 ; espérons que cet arrêt se pérennise. j'aimerais, à partir de quelques exemples concrets, vous démontrer l'impact que la diminution de ces missions peut avoir sur les services offerts à la personne. Je commencerai par la suppression de la compétence de signature des certificats de vie par les consulats. Les Français sont désormais invités à faire signer ces documents par les autorités locales, qui, souvent, refusent parce que le formulaire n'est pas dans la langue locale ou que cet acte ne leur

La suppression de l'accueil téléphonique dans les postes consulaires pose aussi de sérieux problèmes pour les prises de rendez-vous ou d'information, qui ne peuvent se faire que par internet, de nos compatriotes n'ayant pas la faculté Les exemples sont nombreux, mais je n'ai pas le temps, ici, de tous les énumérer. Madame la ministre, je souhaiterais que vous nous indiquiez si de nouvelles missions de service public exercées par les postes consulaires sont appelées à se réduire ou disparaître dans les prochains mois.

Je vais essayer d'apporter une réponse sur plusieurs situations précises que vous avez évoquées. S'agissant des certificats de vie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse prévoit effectivement que les pensionnés doivent se présenter auprès des autorités locales pour faire compléter un certificat de vie. Dans le cas où les autorités locales ne seraient pas fiables

et la compétence notariale des postes consulaires a été restreinte partout où des alternatives locales par des experts compétents s'offraient à nos compatriotes pour un meilleur service.

comme le fait, d'ailleurs, l'ensemble de nos grands partenaires. Cette externalisation permet de concentrer le travail de nos agents sur l'instruction des demandes et la délivrance des visas, soit les étapes à plus forte valeur ajoutée, si je puis m'exprimer ainsi, dans ce traitement des dossiers. possibilité de joindre les consulats par téléphone, plus de 100 000 appels ont été gérés de la mi-mars à la mi-juin par le consulat général de France à Madrid. Ce n'est qu'un exemple, mais il montre tout de même que les permanences téléphoniques existent bien dans nos consulats.

et de l'innovation. Madame la ministre, la bourse au mérite pour les lycéens et l'aide au mérite pour les étudiants sont des aides accordées aux élèves les plus méritants. La première est attribuée après l'obtention d'une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet, et avec l'engagement de poursuivre avec assiduité une scolarité jusqu'au baccalauréat, tandis que la seconde est attribuée après l'obtention d'une mention « très bien » au baccalauréat et l'inscription dans un établissement supérieur. La principale contradiction actuelle réside dans le fait qu'il est nécessaire de bénéficier de la bourse de lycée ou d'une bourse sur critères sociaux pour pouvoir prétendre à la bourse au mérite ou à l'aide au mérite. Pour poursuivre dans les définitions, je vous donnerai, mes chers collègues, celle du terme « mérite », ainsi rédigée dans le dictionnaire Larousse : « ce qui rend quelqu'un (ou sa conduite) digne d'estime, de récompense, eu égard aux difficultés surmontées ». Madame la ministre, la difficulté pour un jeune ou une jeune réside-t-elle nécessairement dans le statut social de ses parents ? Le mérite ne peut-il pas s'illustrer dans le fait, pour un jeune ou une jeune, de surmonter un deuil, le divorce de ses parents, de se diriger vers une voie qui n'était pas souhaitée par son cercle familial ? Plus généralement, le mérite ne consiste-t-il pas, tout simplement, à réussir là où beaucoup échouent, et cela même sans poser la question de l'origine sociale du collégien ou du lycéen, qui, à force de travail, obtient une mention ? À une époque où la classe moyenne éprouve un sentiment grandissant d'injustice en matière de fiscalité, il serait peut-être opportun d'envoyer un signal fort, en permettant à de nombreux élèves et étudiants issus de cette classe sociale de bénéficier de ce dispositif d'aide. En effet, bon nombre de familles sont ostracisées de toutes les aides sociales, alors même qu'elles ne respirent pas l'opulence. Pour toutes ces raisons, madame la ministre, j'aimerais connaître votre position sur une possible modification des règles d'attribution de la bourse et de l'aide au mérite, afin que la notion même de mérite retrouve son sens originel. La parole

Il est passé de 471 000 étudiants en 2007-2008 à 718 000 étudiants en 2019-2020, soit une hausse de 52 %. Cette croissance est supérieure à celle de la population étudiante, où le taux de boursiers est passé de 21 % à 37 %.

62 %. Madame la sénatrice, le double effet de l'élargissement du champ des boursiers et de l'augmentation du nombre de bacheliers obtenant une mention- le taux est passé de 3,2 % à 10,9 % pour la session 2020 -répond à ces objectifs. Vous avez raison : le mérite

en 2010, par un rapport d'inspection favorable à son ajout dans la circulaire Lang et à l'extension de son enseignement. Ce rapport fut aussi élogieux qu'ignoré. La poursuite de cet enseignement est tolérée, mais la continuité pédagogique au collège n'est pas assurée, malgré l'adhésion de 80 % des familles concernées. Au mois de septembre 2019, nous n'avons pu que constater le non-remplacement du seul enseignant de flamand occidental à la suite de son départ à la retraite. À ce jour, aucun enseignant n'a été nommé pour le remplacer. Une délégation menée par le président de l'institut de la langue régionale flamande a été reçue par la rectrice le 11 octobre dernier, dans un climat compréhensif. La reprise d'une expérimentation au lycée et, par voie de conséquence, au collège et à l'école primaire semble en bonne voie. Néanmoins, la non-inscription du flamand occidental dans la circulaire relative aux langues régionales bloque toutes les évolutions de ce dossier, un terreau très favorable : la région des Hauts-de-France soutient la création d'un office public du flamand. Je précise que l'assimilation du flamand occidental au néerlandais n'a pas lieu d'être. Cette conception inique a donné lieu à de nombreux cas de diglossie chez nos amis belges transfrontaliers, apprenant le néerlandais à l'école et parlant le flamand occidental dans leur vie sociale. Dans le Nord, les élèves sont impatients de renouer avec leur héritage culturel et les parents d'élèves sont pressés que l'école de la République accepte les langues régionales comme des réalités. Nous sommes en mesure de proposer des enseignants. Ma question est donc la suivante : allez-vous ajouter le flamand occidental à la liste des langues régionales reprise dans la circulaire

est attaché à la préservation et à la transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des régions françaises. La situation de l'enseignement des langues régionales fait l'objet de la plus grande attention dans les académies et dans les territoires concernés.

au regard de nombreux critères : l'étendue géographique de la zone dans laquelle la langue est pratiquée, la proximité entre le flamand et le néerlandais, reconnue par de nombreux spécialistes de la langue, ainsi que le nombre d'élèves concernés.

un ensemble de 92 élèves volontaires répartis entre trois écoles et trois niveaux de classe, CE2, CM1 et CM2. L'heure hebdomadaire de flamand occidental était incluse dans le volume horaire standard d'enseignement. d'enseignement. Les élèves et les familles n'ont pas souhaité poursuivre cet apprentissage au-delà de l'école élémentaire. Parvenu à son terme, ce cycle d'expérimentation n'a donc pas débouché sur une dynamique de développement permettant la poursuite de l'action. Il est du reste à noter qu'aucune réclamation de parent d'élève ne nous a été communiquée par l'inspecteur de la circonscription. Toutefois, le flamand occidental peut être valorisé par le biais d'autres dispositifs existants. Je pense notamment aux activités éducatives et culturelles complémentaires

des sports. Madame la secrétaire d'État, je me permets de vous interpeller après avoir appris par les maires que les inspections académiques avaient pour consigne de ne plus prendre en charge les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) sur le temps périscolaire. En 2013, les parlementaires votaient la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, où figurait le principe d'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction.

Jean-Michel Blanquer avait eu l'occasion de le rappeler devant la représentation nationale, notamment à la suite d'une question de Mme Françoise Gatel : la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales devait être clarifiée être clarifiée et les décisions du Conseil d'État de 2011, que vous citez dans votre question, ne pouvaient faire jurisprudence, dès lors qu'elles avaient été rendues dans le cadre de référés. Plusieurs pourvois en cassation ont été introduits par les services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, afin d'obtenir du Conseil d'État qu'il tranche définitivement cette question. C'est chose faite depuis le 20 novembre dernier. Le Conseil d'État a ainsi clairement jugé, par une décision de section- cette procédure témoigne de l'importance que la plus haute juridiction administrative a accordée à cette question qu'il appartenait aux collectivités territoriales de prendre en charge l'accompagnement des enfants en situation de handicap dans le cadre des activités périscolaires ou de restauration scolaire qu'elles organisaient.

qui se heurtaient à des refus récurrents des maires d'assumer la prise en charge de ces enfants sur les périodes relevant de leurs compétences, le ministre avait demandé d'accepter de prendre en charge le coût de l'accompagnement dans l'attente de la décision du Conseil d'État.

ont pourtant pris une licence, souvent onéreuse, afin de pratiquer leur discipline. Nombre d'entre eux sont inquiets. La dernière saison s'est terminée prématurément au mois de mars

aux sportifs amateurs, les équipes réserves des clubs professionnels sont privées de championnat et d'entraînement. Leurs joueurs sont pourtant de jeunes espoirs du sport français. Alors que la France accueillera les jeux Olympiques en 2024, la formation de ces talents sportifs en devenir est compromise. Par ailleurs, la distinction opérée entre mineurs et majeurs semble peu pertinente.

En effet, le produit de la licence est versé, non pas à l'association, mais à la fédération à laquelle elle appartient. Je tiens à saluer le plan d'action en faveur du sport, qui apporte un soutien financier nécessaire aux fédérations. Toutefois, les présidents d'association m'ont alertée sur le fait que, pour la plupart des se matérialiserait que lors de la saison suivante. Souvent, le budget de cette année a été bouclé au mois de mars dernier avec les nombreux partenaires publics et privés, mais la crise frappera durement les budgets de la saison prochaine. De nouvelles aides seront alors certainement nécessaires. Madame la secrétaire d'État, nos associations sportives, si riches de leurs bénévoles, sont désormais au bord de l'asphyxie. Humainement, elles assistent à un désengagement de leurs forces vives. Financièrement- vous le savez -, elles sont exsangues. Sportivement, à la veille des jeux Olympiques de 2024, elles craignent un abaissement particulièrement marqué du niveau de nos athlètes, qui ne sont pas tous professionnels. Pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous allez prendre pour desserrer l'étau dans lequel se trouvent les associations sportives ?

par la covid, sur le plan tant sanitaire qu'économique. On le mesure d'ailleurs à la diminution significative du nombre de licenciés. C'est pourquoi nous agissons pour l'avenir du sport, qu'il soit amateur ou professionnel. Le Président de la République a annoncé, il y a deux semaines, un certain nombre de de mesures concrètes en ce sens. D'abord, c'est le retour depuis samedi dernier des mineurs dans les clubs et les associations pour les pratiques de plein air. En outre, puisque ces structures font face à d'importantes

De plus, dès le début de l'année 2021, une aide de 20 millions d'euros issue du plan de relance sera dirigée vers les fédérations sportives

l'activité sportive en plein air des mineurs a repris. Pour les pratiquants adultes, si les conditions sanitaires le permettent, les activités devraient reprendre le 20 janvier prochain, avec des protocoles sanitaires adaptés et renforcés. Enfin, le Président de la République a annoncé que 5 000 postes de service civique seraient fléchés vers le sport

Ce sont ces jeunes que les missions locales accompagnent, afin de les aider à trouver une formation ou un emploi. En tant que présidente de missions locales, je me félicite des dernières annonces du Gouvernement, notamment du plan « 1 jeune, 1 solution », qui a pris en compte cette situation en doublant le nombre de garanties jeunes. Ce dernier sera

la question du financement des missions locales pour la mise en oeuvre des 100 000 garanties jeunes supplémentaires reste à régler définitivement.

Enfin, les missions locales sont majoritairement des associations et leur trésorerie est limitée à trois mois. Le premier versement du financement de l'État a lieu chaque année au mois

Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Agnès Canayer, je connais votre engagement sans faille auprès des missions locales et je tiens à le saluer. Les missions locales sont un maillon essentiel du service public de l'emploi pour repérer, accueillir et accompagner les jeunes les plus en difficulté. Face à la crise, elles sont pleinement mobilisées pour atteindre l'objectif ambitieux du plan « 1 jeune, 1 solution ». objectif, que vous avez décrit avec justesse, est d'accueillir 50 000 jeunes supplémentaires en parcours garantie jeunes et 80 000 jeunes supplémentaires en parcours cette fin, nous avons augmenté la dotation des missions locales de 100 millions d'euros, pour atteindre un total de 472 millions d'euros en 2021. C'est un effort sans sans précédent. Soyez assurée que je veille, avec Élisabeth Borne, à ce que ces crédits soient versés dans les meilleurs délais. Vous le savez, la subvention accordée aux missions locales est globalisée depuis deux ans. Elle n'est plus spécifiquement affectée au financement de l'un ou l'autre de leurs dispositifs. C'était une demande du réseau, qui a été satisfaite par Muriel Pénicaud pour apporter de la visibilité et simplifier les circuits de financement. Nous n'avons évidemment aucune intention de revenir sur Toutefois, pour des raisons de comptabilité budgétaire, nous avons dû artificiellement séparer cette subvention en deux lignes distinctes. Ce fléchage technique est totalement transparent pour les missions locales et nous l'avons partagé avec l'Union nationale des missions locales Enfin, nous devons nous adapter à la nouvelle situation sanitaire et économique. Compte tenu du récent rebond de l'épidémie et afin de ne laisser personne sur le bord de la route, le Gouvernement a décidé, le 26 novembre dernier, de relever son objectif de 50 000 entrées supplémentaires en garantie jeunes. jeunes. Nous proposerons au moins 200 000 parcours en garantie jeunes en 2021. De nouveaux crédits seront rapidement attribués aux missions locales, qui disposeront ainsi de tous les moyens

derrière des démonstrations administratives fumeuses, on a décidé de transférer une part significative des effectifs du commissariat d'Arpajon à celui de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ces commissariats deviennent de simples « antennes de police » et la présence des forces de l'ordre s'en trouve dégradée dans de vastes territoires. Cette réorganisation aura des conséquences néfastes pour la proximité des forces de l'ordre et leur capacité d'intervention au sein de territoires à la démographie dynamique.

et 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires auront été recrutés d'ici à la fin du quinquennat. Pour répondre plus précisément à votre question, les services territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique se réforment- vous l'avez dit -depuis des années, dans une logique de police d'agglomération et de déconcentration, en application de la nouvelle doctrine d'emploi et d'organisation. Il nous est apparu nécessaire de rationaliser les structures et les moyens pour améliorer l'efficacité de l'organisation et mieux répondre aux nécessités opérationnelles. objectif est d'accroître la pertinence de l'architecture territoriale et de dégager du potentiel opérationnel pour une meilleure couverture policière et des capacités d'investigation judiciaire accrues.

Ces maires ne sont qu'en très petit nombre et leur continuité dans ces fonctions traduit, à l'évidence, leur grand dévouement au service de la vie publique ainsi que la qualité exceptionnelle de leur travail, puisque les électeurs leur ont fait constamment confiance. Or si certains d'entre eux ont reçu une distinction honorifique importante, au moins l'ordre national du mérite, ce n'est pas le cas de tous. Quelques-uns ont été oubliés, sans que cette lacune ait aucune justification. Ne faudrait-il pas remédier à cette différence de traitement ? de traitement ? Il ne s'agit pas d'accorder une distinction à l'ancienneté, c'est là le rôle de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale. Il s'agit plutôt de souligner des mérites et un dévouement sur une durée exceptionnellement longue, qui ont été constamment confirmés et reconnus par le corps électoral.

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, mon cher collègue. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable,